d'encadrer encore plus strictement les dispositions relevant de cet hébergement hôtelier, en ne l'autorisant que de façon exceptionnelle et le temps nécessaire à l'évaluation de la situation des demandeurs. Quel est l'avis de la commission

formant un socle en deçà duquel l'accompagnement des enfants et des jeunes majeurs ne pourrait être assuré dans des conditions de sécurité requises, tant pour les enfants que pour les professionnels. Des travaux sont en cours en vue de l'élaboration d'un décret fixant ces normes et critères d'encadrement dans les établissements de la protection de l'enfance. Ils sont néanmoins loin d'être aboutis. Une inscription dans la loi garantirait leur finalisation et leur extension aux services mettant en oeuvre les mesures de milieu

tous personnels confondus. Ce taux varie selon la structure et, s'agissant des catégories de personnel, il existe également des disparités selon les territoires et entre établissements. Comme le relève le Conseil national de la protection de l'enfance dans un avis de novembre 2020, cette situation peut parfois être source de difficultés et de dysfonctionnements. d'établir favoriseraient un traitement équitable des enfants, indépendamment du lieu, des modalités d'accueil et d'accompagnement. Comme l'a rappelé mon collègue Daniel Chasseing, des travaux sont en cours pour élaborer le décret, mais une inscription dans la loi garantirait, selon nous, leur finalisation et leur extension.

de loi transmis au Conseil d'État. Ce dernier a estimé, dans son avis, que ces dispositions étaient déjà satisfaites par le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette base légale s'avère suffisante pour fixer par décret des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement, notamment en matière de taux d'encadrement. Il revient donc au Gouvernement de prendre ces mesures qui, sur le fond, me paraissent très utiles. L'avis est défavorable.

France (ADF). Nous travaillons sur un certain nombre de critères de ressources humaines de base, avec des critères de majoration liés à l'âge des enfants, à la diversification des activités, à la configuration des lieux, à l'architecture du bâtiment.

Ces structures ne sont pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et n'ont pas recours aux financements publics. En effet, il n'y a pas d'organisme « financeur » pour les LVA ; il y a des « utilisateurs », qui paient une prestation de services délivrée par des entreprises de droit privé. Le terme « financement » est donc inapproprié. Nous proposons de revenir à un système de convention bilatérale entre les conseils départementaux et les LVA, permettant d'adapter les conditions de tarification à la réalité de chaque structure et aux prestations spécifiques offertes selon le degré d'exigence de prise en charge. Il sera ainsi possible d'assurer une spécificité à chaque lieu de vie et d'accueil en fonction des besoins.

Ils sont toutefois soumis à une procédure d'autorisation et, leurs « utilisateurs » étant des personnes publiques, il me paraît souhaitable de maintenir un encadrement par décret des modes de tarification. Par ailleurs, notons qu'il est déjà prévu que chaque organisme financeur puisse conclure avec le LVA une convention triennale de prise en charge, déterminant notamment les conditions d'exercice des prestations et les modalités de versement des forfaits journaliers.

examiner de près le cahier des charges, le nombre de personnes qui interviennent, la qualité de l'accueil, de l'accompagnement, l'environnement des jeunes, les activités extérieures. C'est un travail qui demande beaucoup de temps,

secrétaire d'État. Je l'ai évoqué dans la discussion générale, les députés ont inscrit pour la première fois dans le code de l'action sociale et des familles le principe du parrainage. Je vous suggère d'aller plus loin, et ce à double titre.

En France, près de 1 000 enfants sont aujourd'hui accompagnés par le réseau France parrainage. Nous nous réjouissons que ce dispositif soit consacré dans la loi et renforcé par l'amendement que nous venons de voter, tant il démontre son utilité en offrant aux mineurs un soutien affectif et éducatif d'une grande importance, ainsi qu'une ouverture sociale et culturelle, une échappatoire au cadre existant, un soutien dans les moments difficiles, autant d'éléments essentiels à l'accompagnement vers l'autonomie. Toutefois, un élément essentiel manque au dispositif tel qu'il est présenté dans ce projet de loi, à savoir le fait d'inscrire ce projet de parrainage au sein du projet pour l'enfant Or cela fragilise le dispositif du parrainage puisque, n'étant pas inscrit dans le PPE de l'enfant, le lien privilégié que le dispositif tend à construire peut être rompu en fonction de l'évolution administrative de la situation de l'enfant. Nous devons, au contraire, renforcer le dispositif en l'inscrivant dans le projet pour l'enfant afin de préserver et de stabiliser le lien que le dispositif construit. Cela aura pour bénéfice, par ailleurs, de lever un peu plus les freins au développement de ce dispositif, partout en France. Par le biais de cet amendement, de renforcer le dispositif que nous saluons par ailleurs. Quel est l'avis de la commission ? Notre collègue propose que le projet de l'enfant évalue l'opportunité de mobiliser la société civile pour les enfants protégés à travers une relation de parrainage. Cet

En 2019, la députée Perrine Goulet, écrivait dans un rapport d'information sur l'aide sociale à l'enfance que l'ampleur des problèmes sociaux rencontrés dans certains établissements de l'ASE justifiait la mise en place d'une véritable politique nationale de contrôle.

Nombre d'articles, de travaux, d'investigations, de documentaires, de livres, de témoignages font état de violences dans certaines familles ou dans certains centres de l'ASE.

de la députée Florence Provendier. L'actualité récente a mis en lumière des dysfonctionnements particulièrement graves de certains établissements de la protection de l'enfance. Il semble nécessaire, par conséquent, d'autoriser sans restriction l'accès des parlementaires aux établissements de l'aide sociale à l'enfance, raison pour laquelle nous soutenons l'idée de créer un droit de visite de ces établissements, sur le modèle du droit de visite des lieux de privation de liberté. Quel

le contrôle en revient au département. Ce qui se passe au domicile, y compris de gré à gré, avec des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées, personne ne peut le vérifier, pas même l'inspection du travail. C'est ainsi, c'est le domicile

Cet article amorce une politique de prévention des sorties sèches qui nous semble insuffisante pour réduire la surreprésentation massive des jeunes étant passés par l'aide sociale à l'enfance dans la précarité économique et résidentielle par rapport à leur catégorie d'âge. Combien de temps allons-nous encore exiger de ces jeunes, dont le parcours est marqué par de nombreuses ruptures, séparations, une faiblesse d'entourage familial et amical, les mêmes gages dans

L'exigence d'autonomie est beaucoup plus forte et plus précoce à l'égard des jeunes protégés que pour la population des jeunes en général. » L'âge de la majorité représente en effet un couperet contre-productif qui sape le travail d'insertion sociale de l'ASE. Rappelons que la fonction de l'ASE est celle d'une suppléance parentale. Alors que l'âge moyen de décohabitation des jeunes est de 25 ans et que leur premier emploi stable est obtenu à 27 ans, les parcours et les caractéristiques des jeunes placés, y compris en termes de santé et de niveau de qualification,

L'insertion du majeur issu de l'aide sociale à l'enfance nécessite que, dès sa prise en charge par les services de protection de l'enfance, des politiques de long terme soient mises en oeuvre. La protection de l'enfance en ce sens joue un rôle central dans le développement des mineurs et dans leur insertion, tant dans le dispositif qu'une fois qu'ils en sont sortis à leur majorité. commission ? Cet amendement vise à ajouter au sein des missions de la protection de l'enfance celle de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de l'enfant. Cette précision présente une portée pratique assez limitée : l'insertion professionnelle

engagé depuis trois ans au moins sur la question des sorties de l'aide sociale à l'enfance, notamment les sorties sèches. Une étude récente de la direction générale de la cohésion sociale monte que 57 % uniquement des enfants bénéficient toujours d'un accompagnement une fois qu'ils ont passé l'âge de 18 ans. Ces chiffres ont été rappelés à plusieurs reprises un sans domicile fixe né en France sur quatre est passé à un moment ou à un autre par l'aide sociale à l'enfance. Il existe par ailleurs de grandes inégalités territoriales d'un département à l'autre sur la poursuite de l'accompagnement à la majorité. en place de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, l'État, en responsabilité, et parce que l'insertion professionnelle, monsieur le sénateur, est au coeur de ses compétences,

Sénat : la référence à des difficultés d'insertion sociale, lesquelles étaient une des conditions pour mettre en place l'accompagnement. Là aussi, nous avons supprimé cette notion.

l'amendement n° 387. Le Défenseur des droits rappelle, dans sa décision du 27 décembre 2018, que les juridictions administratives ont jugé à plusieurs reprises que la durée de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ne constituait pas en soi une motivation suffisante de refus d'une prestation d'accueil en faveur d'un jeune majeur. Au contraire, comme l'a confirmé la cour administrative d'appel de Nantes, les difficultés d'insertion d'un jeune majeur peuvent au demeurant être accrues par l'absence ou la durée limitée de prise en charge en qualité de mineur. Actuellement, la loi ne subordonne pas l'accès à une prise en charge jeune majeur au fait d'avoir été confié en tant que mineur à l'ASE. Cependant, les départements ont émis des règlements qui posent déjà cette condition, en prévoyant parfois une exigence de durée minimale de prise en charge durant la minorité. Le Conseil d'État a dû se prononcer à plusieurs reprises pour rappeler que les conseils départementaux ne peuvent fixer de nouvelles conditions conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ de la loi. Ces pratiques risquent, selon l'Unicef, de trouver une base légale et d'être amplifiées avec cette rédaction de l'article 3 D. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cette condition afin de permettre l'accompagnement des jeunes majeurs confiés ou non à l'aide sociale à l'enfance durant leur minorité. La parole

Apourceau-Poly. Chaque jeune de moins de 21 ans qui sort du dispositif de la protection de l'enfance doit être accompagné par l'État ou par le département. Actuellement, 64 % des départements conditionnent l'attribution d'un accueil provisoire jeune majeur à une prise en charge antérieure par l'ASE, avec des critères de durée plus ou moins restrictifs. Ces critères restrictifs correspondent à un alignement des aides par rapport aux dotations des départements pour la protection de l'enfance. Il faudrait donc, selon nous, inverser la logique et adapter les aides aux besoins des jeunes majeurs. Dans la situation actuelle, cela signifie qu'au moins 64 % des départements ne proposent pas de solution aux jeunes majeurs qui n'ont pas été confiés à l'ASE avant leur majorité, ce qui est complètement injuste. Pour ces raisons, nous souhaitons, par cet amendement de repli, généraliser à l'ensemble des jeunes majeurs de moins de 21 ans une prise en charge à titre temporaire, même s'ils n'ont pas été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité. Quel

Les confinements successifs ont rendu visible une problématique ancienne, celle du rejet, de la violence, et parfois de la haine, dont peuvent faire l'objet les jeunes LGBTI au sein même du cercle familial,

Les signalements au sein de la famille sont en constante augmentation. Aujourd'hui, c'est le secteur associatif qui accueille les jeunes LGBTI. Ces associations font un travail incroyable et nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Cet amendement prévoit une mesure simple, c'est-à-dire de moins de 21 ans puissent être protégés et accueillis par l'aide sociale à l'enfance, car il est plus que temps que l'accueil des jeunes LGBTI en situation de détresse soit une politique publique assumée par l'État, plutôt qu'une politique sous-traitée aux associations.

la promulgation de la présente loi, sur l'opportunité de la systématisation de l'accompagnement des jeunes majeurs pris en charge par l'ASE jusqu'à l'âge de 21 ans. Une proposition de loi de nos collègues députés socialistes vient d'être déposée en faveur de l'accompagnement jusqu'à 25 ans des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort en effet d'une étude de la Drees que l'âge moyen de départ du foyer parental en 2018 était de 23,7 ans, et de 26 ans pour l'ensemble des jeunes européens. Les jeunes qui sortent de placement doivent accéder à l'autonomie et à l'indépendance beaucoup plus tôt que les autres. Leur chemin vers l'âge adulte est bousculé et accéléré, alors qu'ils cumulent les difficultés sociales et familiales. Les chercheurs en sciences sociales constatent en effet qu'une grande partie de ces jeunes connaît un retard scolaire, un plus faible niveau de diplôme, de plus grandes probabilités de rencontrer des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, de parentalité précoce, de délinquance ; ils risquent aussi d'entrer rapidement sur le marché du travail dans des emplois précaires et peu rémunérés. Un quart des jeunes en fin de parcours à l'ASE sont en rupture de liens parentaux, soit parce qu'ils sont orphelins des deux parents, soit parce qu'ils ont subi une rupture précoce de leurs liens avec leurs parents, à la naissance ou durant leur parcours de de placement. En plus de vivre des difficultés socioéconomiques, leur isolement est donc central. Le prolongement de l'aide aux jeunes majeurs constitue alors un levier pour les accompagner dans leur passage à l'âge adulte. Quel est l'avis de la commission ? Comme

de veiller à l'accès et à la continuité des soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. Nous le savons, un quart des enfants placés sont en situation de handicap. Comme tous les enfants pris en charge par l'ASE, ils doivent pouvoir

nationale. Cet article avait pour objet d'intégrer au rapport annuel pourtant sur la situation des mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance un bilan pédiatrique, psychique et social.

Le fait que cet article consacre désormais dans le code civil l'existence de ces dispositifs renforcés et de cet accompagnement spécialisé est une avancée. Cet accompagnement peut être long et se heurter à des situations complexes qui prennent du temps à être déconstruites et dénouées. La durée d'une mesure d'assistance doit pouvoir varier et s'adapter à chaque situation particulière de l'enfant. C'est au juge des enfants qu'incombe la responsabilité d'évaluer la situation et de délimiter le temps de l'assistance en tenant compte de la gravité de la situation. Aussi, délimiter si strictement le temps de ces actions éducatives alourdit le travail des juges, alors même que le temps défini est parfois trop court. Le Syndicat de la magistrature relève que les AEMO renforcées de six mois sont, en pratique, très souvent insuffisantes. Cet amendement vise donc à supprimer la limitation de six mois en rendant au juge son pouvoir d'appréciation et en lui laissant la possibilité de définir des AEMO plus adaptées à la particularité de chaque situation.

fixe la durée de la mesure, sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut par ailleurs être renouvelée par décision motivée. En outre, il semblerait que les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert de six mois soient parfois insuffisantes, ce qui obligerait le juge à réexaminer la situation.

au rétablissement de la rédaction initiale de l'Assemblée nationale, qui introduisait la possibilité pour le juge des enfants d'ordonner une mesure de médiation familiale en complément d'une mesure d'assistance éducative. En effet, en commission des affaires sociales du Sénat, cette disposition a été complétée par la précision les parents devront être informés par le juge des enfants des mesures d'aide éducative dont ils pourraient bénéficier dans un cadre administratif. Or cette information est déjà donnée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, en application de l'article L. 223-1 du code de l'action sociale et des familles. Il ne nous semble pas nécessaire

et donc hors du cadre de la médiation familiale ordonnée par le juge. Les informations relatives à cette protection doivent donc être délivrées aux parents par le conseil départemental qui en a la charge, et non par le juge des enfants. problème de coordination. Pour toutes ces raisons, il convient, nous semble-t-il, de revenir à la rédaction suivante : « Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées

On retrouve ici des difficultés précédemment pointées dans les textes sur les violences intrafamiliales. Comment qualifier ou repérer l'emprise de manière manifeste ? De même, on sait que des mères victimes de violences conjugales peuvent, par peur, chercher à tout prix à dissimuler les violences dont elles sont victimes ou les nier. Dans les situations de violences intrafamiliales, la médiation, qu'elle soit pénale ou familiale, est déconseillée en toutes circonstances. Pourtant, il a fallu de nombreux efforts aux associations spécialisées, aux avocats et aux militants des droits des femmes pour obtenir par voie législative l'interdiction formelle de la médiation familiale dans les situations de violence conjugale. La circonspection est donc de mise. Même s'il est utile et opportun d'aider les parents à résoudre des différends familiaux qui ne sont pas source de violence, il est important que cette médiation familiale soit conditionnée à l'audition préalable de chacun des parents, séparément, et de leurs enfants. Quel l'avis de la commission ? recueillir l'accord des parents pour cette désignation, ce qui pourra nécessiter des auditions séparées. Il me semble donc préférable de laisser au juge le soin d'apprécier, selon chaque situation, les modalités d'entretien qui lui paraissent adaptées, sans prévoir systématiquement un entretien obligatoire au risque de surcharger le cabinet du juge, qui pourrait alors être désincité à proposer cette mesure. il serait peu opportun d'obliger le juge à entendre tous les enfants, même ceux qui ne sont pas capables de discernement, pour cette seule mesure de médiation, alors que ce n'est pas obligatoire pour les autres procédures. Enfin, la réalisation d'entretiens individuels sera par la suite la mission du médiateur qui sera désigné. L'avis est donc défavorable.

de fluidifier les relations et de permettre un traitement facilité, voire une résolution plus rapide, des situations d'enfants à la fois porteurs de handicap

le Défenseur des droits a publié un rapport sur le handicap et la protection de l'enfance. Les données recueillies font état d'un taux de prévalence du handicap sept fois supérieur parmi les enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par rapport à la population générale. sur les statistiques : près de 70 000 enfants seraient en situation de handicap sur les 308 000 enfants faisant l'objet d'une mesure d'aide sociale. L'IGAS, dans un rapport de 2011, évaluait la prévalence des handicaps seulement psychiques à 25 % des enfants pris en charge par l'ASE, ce que confirme le Défenseur des droits. Le handicap chez les enfants suivis par la protection de l'enfance est donc une problématique majeure, qui n'est pas traitée par ce projet de loi. la raison pour laquelle la désignation au sein de chaque conseil départemental et de chaque maison départementale des personnes handicapées d'un référent institutionnel permettrait un traitement facilité, voire une résolution plus rapide, des situations d'enfants à la fois porteurs de handicap et relevant de la protection de l'enfance. La mise en place de ce référent, qui n'est pas encore effective, pourrait permettre une meilleure coordination entre les organisations et les acteurs impliqués, le Défenseur des droits dénonçant à ce sujet une gouvernance émiettée et illisible.

l'amendement n° 146. Nous avons déjà évoqué les énormes difficultés d'insertion des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Le constat est sans appel

introduit à l'Assemblée nationale, permettant l'accès des jeunes sortant de l'ASE au dispositif du logement social en tant que public prioritaire. Il s'agit d'une mesure de bon sens qui vise à réduire l'inégalité de fait devant le droit au logement, condition essentielle de l'insertion sociale et professionnelle

mais une manière de la diminuer est d'entamer une politique du logement à la hauteur des besoins plutôt que de renoncer à établir une liste de publics super-prioritaires au regard des urgences sociales. Les personnes en grande précarité et en grande pauvreté sont des victimes

C'est pour cette raison que notre amendement rétablit l'article modifiant le code de la construction et de l'habitation, afin de permettre aux jeunes majeurs qui sortent du dispositif de protection de l'enfance et qui ne sont pas étudiants de bénéficier de manière prioritaire d'un logement social.

une stabilité résidentielle pour plus de sérénité et moins de précarité. Pour cela, nous le savons tous, le parc social joue un rôle central. Les logements, plus accessibles financièrement que ceux du marché privé, sont la clé pour garantir une stabilité résidentielle, la durée du bail étant illimitée. étant illimitée. Toujours dans le but de renforcer l'insertion des jeunes majeurs et de leur proposer des solutions concrètes pour répondre aux difficultés auxquelles ils peuvent faire face, nous souhaitons rétablir le dispositif permettant aux jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance de bénéficier d'un logement social de manière prioritaire. La parole

Les arguments avancés par le rapporteur pour justifier le fait que les jeunes majeurs suivis par l'ASE ne soient pas prioritaires pour l'attribution d'un logement social ne sont pas recevables. Certes, la liste des publics prioritaires, comprenant par exemple les personnes victimes de violences conjugales, les personnes sortant de la prostitution, ou celles en situation de handicap, Mais pourquoi ne pas également y inclure les jeunes majeurs suivis par l'ASE ? Monsieur le rapporteur, vous dites que ces personnes entrent déjà bien souvent dans ces critères. Les difficultés sont en effet généralement cumulatives, mais ceci est également valable pour les critères déjà existants : une personne handicapée peut aussi être victime de violences, ou rencontrer des difficultés financières ou d'insertion sociale. Quant à votre argument selon lequel en introduisant cette catégorie supplémentaire on risquerait de retarder encore plus l'accès au logement social faute de logements suffisants, ce n'est pas sérieux

Dans le Val-de-Marne, la ville de Saint-Maur-des-Fossés ne compte que 8,3 % de logements sociaux et Saint-Mandé 10,8 %. La solidarité et l'accompagnement des personnes les plus vulnérables ne font pas partie de vos priorités.

que l'entretien de préparation à l'autonomie soit effectué au plus tard un an avant la majorité du mineur pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. La Défenseure des droits s'est inquiétée de cette disposition du fait que de nombreux mineurs- notamment des MNA -sont pris en charge après l'anniversaire de leurs 17 ans. Si l'entretien de préparation devait être réalisé avant leur entrée dans le dispositif, ces mineurs en perdraient le bénéfice.

suggéré par l'association Repairs ! vise à compléter l'alinéa 4 pour renforcer l'accompagnement d'un jeune lors de l'entretien avec les services de l'ASE un an avant sa majorité.

Les responsables de l'association Repairs ! nous expliquaient qu'il était très anxiogène pour ces jeunes de n'avoir aucune visibilité sur les soutiens dont ils peuvent bénéficier après leurs 18 ans. Cet amendement oblige ainsi les services départementaux à explorer ces possibilités, et à informer les mineurs un an avant leur majorité. Nous avons bien suivi les débats à l'Assemblée nationale sur cet amendement, qui pour nous a un objet situé bien au-delà de la notification des droits. L'un des enjeux de la protection de l'enfance est précisément

qui évoquait les missions locales, qu'un accord a été passé entre l'Assemblée des départements de France, la Cnape et l'Union nationale des missions locales, pour que les missions locales soient davantage investies dans l'accompagnement vers l'insertion professionnelle des jeunes. Nous savons que des disparités nationales existent, et que toutes les missions locales ne se valent pas. C'est une réalité. Mais toutes doivent désormais identifier le public de l'aide sociale à l'enfance comme l'un des publics prioritaires dans l'accompagnement

dès lors de rappeler que ce projet d'accompagnement doit être envisagé avec le jeune, dans un esprit de coconstruction. L'amendement n° 209 rectifié n'est pas soutenu.

former un recours à l'encontre de la décision prise, conformément à leurs droits. Néanmoins, la rédaction actuelle du projet de loi pourrait laisser penser que le projet d'accompagnement est présenté au jeune concerné sans que ce dernier ait été impliqué dans son élaboration. Il importe dès lors de rappeler

3 instaure un entretien postérieur à la majorité pour dresser le bilan du parcours et de l'accès à l'autonomie du jeune majeur. Néanmoins, aucun accompagnement n'est réellement prévu afin de rechercher des solutions alternatives et effectives, ce qui a alerté la Défenseure des droits.

qui prévoit qu'une des missions de cet entretien est de faire le bilan de l'accès à l'autonomie du jeune. Le service de l'ASE peut donc communiquer au jeune les informations sur les solutions qui s'offrent à lui.

stigmatisation ni harcèlement. Quel

187 000 mineurs et jeunes majeurs étaient pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Leur placement est motivé par la nécessité de les protéger de la violence familiale, de pallier la défaillance ou l'absence des parents. Dans le cadre d'une enquête sur l'accès à l'autonomie de ces jeunes, des journalistes du quotidien ont réalisé des entretiens auprès d'une centaine d'entre eux au cours de la période qui suivait leur sortie de placement. Lors de ces échanges, environ un jeune sur trois a évoqué de façon spontanée des faits s'apparentant à de la violence lors du placement. Ce n'est pas la majorité, fort heureusement, mais, nous le savons, ces faits existent. Les témoignages laissent apparaître deux grandes catégories de violences : celles survenant dans les interactions personnelles que les jeunes ont au quotidien, et celles qui sont liées aux politiques publiques et au fonctionnement de l'institution. La violence est plus souvent psychologique que physique, et passe par la dévalorisation, le dénigrement, le manque d'affection.

Il est donc indispensable que les missions de l'aide sociale à l'enfance soient accomplies sans violence physique ou psychologique sur l'enfant, conformément aux avis rendus par le Défenseur des droits et Unicef France. Quel

est à M. Xavier Iacovelli. Cet amendement a pour objet le renforcement du contrôle réalisé par l'aide sociale à l'enfance sur les conditions de placement des mineurs protégés.

cette raison, nous proposons de compléter ces dispositions pour renforcer le contrôle effectué par les services à travers le prisme de la qualité des conditions d'accueil que nous souhaitons voir explicitement mentionnée dans cet article. Nous constatons en effet que les contrôles actuels ne permettent pas de prévenir au mieux les situations de maltraitance et doivent absolument être approfondis pour lutter efficacement contre ces situations mettant en péril la sécurité des enfants concernés. Quel est l'avis de la commission ? Monsieur Iacovelli, vous avez raison : il faut absolument contrôler les établissements beaucoup plus fortement que l'on ne le fait.

et un sans-abri sur quatre est issu de l'ASE. Il paraît essentiel de renforcer l'accompagnement vers l'autonomie des jeunes majeurs issus de l'ASE, jusqu'à ce qu'ils obtiennent un emploi stable et, au plus tard, jusqu'à 25 ans. C'est une possibilité qui est donnée aux départements.

et personne ne propose de limiter ces dispositifs familiaux à la majorité des enfants. Et pourtant, les autorités publiques, qui assurent une responsabilité de suppléance parentale, ne s'obligent pas au même soutien. De la Défenseure des droits à la Cour des comptes, tous soulignent l'absurdité du système d'accompagnement des jeunes sortis de l'ASE, même si cette loi l'améliore effectivement concernant les sorties sèches. nous nous accommodons de demi-mesures, qui produisent de la précarité, de la pauvreté, du « sans-abrisme » chez les jeunes qui pourtant nous ont été confiés. Il faut aller plus loin, plus fort. cette raison, nous proposons de prolonger la possibilité d'une prise en charge des jeunes majeurs par les services de protection de l'enfance jusqu'à l'âge de 25 ans, soit l'âge moyen de la décohabitation,

refusée. Nous proposons une mesure de justice sociale en faveur d'un public marqué par beaucoup d'épreuves. La parole

à l'ASE. En réalité, l'accompagnement jusqu'à 25 ans est déjà pratiqué par certains départements. Dans la mesure où la loi n'interdit pas de continuer la prise en charge jusqu'à cet âge si la situation du jeune le nécessite, je vous propose de ne pas adopter cette mesure. En outre,

Le présent amendement vise à permettre aux mineurs et aux jeunes majeurs pris en charge ou antérieurement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'aux personnes adoptées qui recherchent leurs origines, de bénéficier de l'accompagnement systématique, lors de la lecture de leur dossier, de travailleurs sociaux

code civil pour établir,, qu'un mineur qui se prostitue doit être considéré comme victime. La question du consentement continue de se poser dans des cas de prostitution,

prévu à l'article 226-13 du code pénal. Il s'agit d'étendre le dispositif de levée du secret professionnel dès lors qu'un mineur exerce une activité prostitutionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ce mineur soit victime de sévices de privations laissant présumer des violences à son encontre. Cette rédaction reprend ainsi les dispositions de l'article 13 de la loi précitée du 4 mars 2002, selon lequel « tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger

par la lecture combinée de l'article 226-14 du code pénal, dont le 2° concerne déjà les mineurs en danger ou risquant de l'être,

cet article est formulé dans des termes généraux, globaux : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises,

à clarifier le régime juridique de l'incapacité d'une personne à intervenir ou à exercer une fonction dans un établissement relevant du code de l'action sociale et des familles en raison de ses antécédents judiciaires. Nous abordons ici la question

atteinte aux personnes et atteinte aux biens -et, d'autre part, à la mention du quantum de la peine prononcée selon le type de délit. Cet amendement tend par ailleurs à modifier l'état du droit en ajoutant les crimes et délits suivants : les destructions, dégradations et détériorations dangereuses, les actes de terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Dès lors que le texte prévoit la consultation du Fijais, il convient de préciser que toute condamnation définitive figurant dans ce fichier entraîne l'incapacité prévue par les nouvelles dispositions, même si la condamnation ne figure plus au bulletin n° 2 du casier

d'exercer une activité professionnelle ou bénévole dans le secteur social et médico-social, en cas de condamnation pour crime ou pour certains délits. Je constate avec satisfaction que le dispositif de l'amendement reprend les apports de la commission, qui a prévu explicitement la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du Fijais pour contrôler les incapacités. Cet ajout procède d'une recommandation de la mission commune d'information sur la répression de violences sexuelles sur mineurs, qui a rendu son rapport en 2019. L'application de ces mesures est indispensable pour assurer une prévention efficace des risques de maltraitance dans les établissements sociaux, qui accueillent des personnes souvent très vulnérables. les contrôles sont peu effectués et cela varie beaucoup d'un secteur à l'autre, d'un territoire à un autre ; cela n'est pas acceptable. Au-delà de l'écriture de la loi, le Gouvernement est responsable de l'application de celle-ci. Je sais que des travaux sont en cours pour déployer

Cet amendement a pour objet de mentionner explicitement la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants dans la politique de prévention ainsi que dans la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance. Il s'agit d'une proposition de

précisant les modalités de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance. Quel est l'avis de

comme un volet complémentaire de la stratégie des établissements de l'aide sociale à l'enfance. Les professionnels exerçant dans ces établissements souhaitent que la santé, prise en compte dans sa globalité, c'est-à-dire intégrant le bien-être des mineurs, soit une priorité de la politique de protection de l'enfance. Pour sa part, la Haute Autorité de santé définit des recommandations qui « prennent en considération la notion de développement et de bien-être, conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant et à la loi [ ...] du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Elles intègrent la santé des mineurs/jeunes majeurs dans la démarche d'accompagnement global et comme comme faisant pleinement partie du projet pour l'enfant. » La prise en compte de la santé globale de l'enfant trouve donc toute sa place dans la stratégie de prévention et de lutte contre la maltraitance Elle ne pourra cependant pas faire l'économie de la formation des professionnels à la prise en compte de la santé en termes de prévention primaire et secondaire, secondaire, d'éducation et de promotion de la santé, ainsi qu'aux besoins du mineur ou du jeune majeur, à la connaissance des problématiques de santé et au repérage précoce des signes d'alertes. commission ? L'amendement me paraît satisfait, dans la mesure où les schémas d'organisation sociale et médico-sociale doivent déjà apprécier les besoins sociaux et médico-sociaux de la population et dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante. J'indique par ailleurs que le pilotage de la santé publique est renforcé à l'article 12 par la définition de priorités pluriannuelles d'action en matière de PMI et que la gouvernance territoriale proposée à l'article 13 , qui sera transversale, permettra aussi d'aborder des questions de santé de l'enfant protégé. La commission est donc défavorable

précise que la stratégie de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en place par les établissements et services de l'aide sociale à l'enfance prévoit un dispositif particulier de prévention et de lutte contre la prostitution des mineurs. Une sensibilisation particulière au risque de prostitution des enfants de l'ASE est nécessaire dans ces établissements, à la fois pour les professionnels en charge des enfants et pour les enfants accompagnés par l'ASE. Il conviendrait de prévoir des réunions associant associant l'ensemble des acteurs, en vue de lutter contre la prostitution des mineurs, de davantage sensibiliser et informer les professionnels dans le cadre de leur formation sur l'existence des réseaux de prostitution, leurs modes de recrutement, les signes d'alerte de développer des partenariats avec les associations spécialisées. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement semble déjà satisfait et peu opportun. Le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, qui devra comporter une stratégie de lutte contre la maltraitance dans les établissements de l'ASE, pourra déjà aborder le sujet spécifique de la lutte contre la prostitution des mineurs, sans qu'il soit besoin de le spécifier dans la loi. Pourront être identifiés des parcours de prises en charge pour ces jeunes entre les différents acteurs. telle précision dans la loi, il faudrait le faire pour de nombreux autres publics spécifiques, qui pourraient être aussi visés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale. Par ailleurs, ces schémas restent centrés sur les établissements sociaux, alors qu'un plan exhaustif et complet de lutte contre la prostitution des mineurs devrait également, pour être transversal et efficace, associer d'autres acteurs tels que les magistrats, les forces de sécurité intérieure et les professionnels de santé.

L'article 5 prévoit que le président du conseil départemental présente à l'assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion des établissements et sur les événements indésirables graves. Cet amendement vise à introduire dans ce rapport le nombre de jeunes suivis par l'aide sociale à l'enfance, par tranches d'âge. Ces données sont déjà collectées par les départements et elles peuvent être agrégées et mises à disposition

doit être nécessairement structurée par une référence nationale commune à tous les acteurs concernés par l'alerte, le repérage et le traitement des risques et des situations de maltraitance. telle définition, permettant de mieux appréhender les phénomènes complexes de maltraitance, est issue du vocabulaire partagé de la maltraitance, transversal aux publics mineurs et majeurs. Elle a été élaborée dans le cadre d'une démarche nationale de consensus menée de 2019 à 2021

Elle sera également inscrite au sein du futur référentiel d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2022. Ce vocabulaire partagé introduit également une caractérisation des différentes situations de maltraitance possibles, pour aider les professionnels et le grand public, en particulier les personnes en situation de vulnérabilité, dans l'analyse collective, la cessation et la prévention des maltraitances.

référence au sein du titre I du livre I du code de l'action sociale et des familles, cette référence commune devient l'un des principes généraux guidant l'action sociale et médico-sociale. Elle permettra de consacrer la politique de prévention de la maltraitance, de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance comme constitutive de cette dernière.

Il est peu probable que cela assure réellement sa diffusion et son application par tous les professionnels. Ces dispositions relèvent effectivement du contenu d'un référentiel, élaboré par la HAS ou par la Commission pour la lutte contre la maltraitance, qui devrait être diffusé aux professionnels en complément de formations et de sensibilisations.

La séance est levée.